et Républicain. Madame la Première ministre, nous nous sommes rencontrés pour la première fois, sur votre demande, le 27 juillet dernier. Je vous avais alors fait part de ma grande préoccupation quant à la situation sociale de la rentrée de septembre et vous avais proposé une revalorisation significative du Smic ainsi que l'organisation d'une grande conférence salariale, afin d'anticiper les difficultés financières prévisibles pour l'immense majorité de nos concitoyens. Vous m'aviez répondu que tel ne serait pas votre choix et que vous privilégieriez la solution des accords de branche. Aujourd'hui, le désordre s'installe, la colère gronde et les premières victimes de cette situation sont les salariés obligés d'utiliser leur voiture. La crise des carburants que traverse notre pays constitue le premier étage d'une crise sociale généralisée installée sur son pas de tir. Les inégalités se creusent et ce n'est qu'un début ... Faire preuve d'autoritarisme en réquisitionnant les salariés sans responsabiliser les employeurs ne permettra pas de revenir à la paix sociale à laquelle nous aspirons Aucune prime, même dite « Macron », limitée dans le temps et dans l'espace, ne remplacera une revalorisation durable des salaires. Vous n'anticipez plus. Vous ne faites plus que corriger, et mal, au moyen de rustines extrêmement coûteuses pour la solidarité nationale, que vous convoquez pour mieux exonérer les plus aisés de nos concitoyens. Les pompes à essence s'assèchent, le pouvoir d'achat est siphonné par l'inflation, mais les dividendes, eux, continuent de ruisseler. Madame la Première ministre, cette situation est absurde certaines entreprises peuvent tripler leurs bénéfices en profitant de la crise actuelle, sans pour autant augmenter leurs salariés, sans contribuer à l'effort national. Ma question est donc simple : face à cette aberration, allez-vous choisir le camp de la résignation ou celui du combat pour la justice sociale ?

Or tous me disent la même chose : les Français veulent vivre de leur travail. Cette conviction, c'est aussi la mienne et c'est celle de mon gouvernement ; le travail, c'est la dignité, c'est l'émancipation. Et c'est bien pour protéger le pouvoir d'achat des Français que nous avons pris des mesures fortes. Je pense notamment au bouclier tarifaire, mesure la plus protectrice d'Europe. depuis plus de cinq ans, nous agissons pour que le travail paye toujours mieux. Je pense notamment à la suppression de certaines cotisations sociales

patron, M. Pouyanné, a augmenté de 52 % son salaire en 2021 afin d'atteindre 500 000 euros par mois ? Voilà ce qui est injuste et que vous ne combattez pas ! Vous êtes faible avec les forts et forte avec les faibles

Monsieur le ministre, les Français vivent depuis maintenant plus de deux ans dans un contexte particulièrement anxiogène, enchaînant crise sanitaire, crise économique, guerre en Europe et inflation générale, tout cela avec une remarquable capacité de résilience, qu'il est important de souligner. s'expliquant par les grèves dans les raffineries, mais également par une augmentation mal anticipée de la consommation liée aux remises à la pompe, est venue donner le coup de grâce à une partie de la population, qui ressent particulièrement la fracture sociale et territoriale des Français qui n'ont aucun accès aux transports en commun et qui n'ont d'autre moyen de locomotion que la voiture. Bien sûr, il y a eu des comportements irresponsables de la part de certains

et c'est avec elle que l'État doit composer : les stations-service sont prises d'assaut, les Français sont confrontés à des difficultés pour se déplacer et des professionnels ne peuvent plus travailler correctement, y compris dans les services essentiels à la population. Je sais que ce n'est pas au Gouvernement de discuter des salaires des grévistes- en tout cas, il n'est pas l'acteur principal de ces négociations -, mais il s'agit ici d'évoquer les problèmes d'approvisionnement relatifs à un bien stratégique qui pourraient potentiellement paralyser jusqu'aux services de santé et de sécurité de notre pays. L'État a donc l'obligation de s'en mêler. Après avoir pris quelques mesures, malheureusement insuffisantes, vous avez annoncé hier que les préfectures pourraient réquisitionner les salariés de certaines raffineries en grève. Pouvez-vous nous préciser comment cette réquisition se déroulera ? Ne craignez-vous pas que la justice vous oppose la liberté fondamentale du droit de grève, comme cela s'est déjà produit en 2010 ? Si tel était le cas, quelles autres pistes pourriez-vous envisager, tout en évitant d'importer davantage de gazole russe, afin de répondre à la demande ?

agit là où il le peut et là où il le doit, depuis le début de cette crise sociale, qui conduit à des situations de tension réelle dans de nombreux départements de notre pays et qui pénalise des millions de nos concitoyens pour se rendre à leur travail, faire leurs courses, amener leurs enfants à l'école, voire, vous l'avez dit vous-même, se soigner. Nous avons d'abord suppléé le carburant qui ne pouvait pas sortir des centres de dépôt en important massivement, notamment depuis la Belgique, du carburant à destination de la région des Hauts-de-France. Nous avons également puisé dans nos réserves stratégiques de carburant et multiplié le recours à des camions-citernes dans une noria organisée de manière à remédier aux difficultés rencontrées par de nombreuses stations-service. Néanmoins, nous avons conscience que cela ne suffit pas à régler le problème.

Cet accord n'a pas été respecté ni soutenu par la CGT, qui a annoncé souhaiter continuer le blocage. L'État prend alors ses responsabilités en demandant au préfet de prendre, dans les plus brefs délais, des arrêtés de réquisition, qui devraient être opérationnels aujourd'hui, de manière à débloquer l'accès au dépôt

semblent avoir décidé de participer aux premières réunions. Nous restons extrêmement attentifs à l'évolution de ces discussions et aux décisions d'arrêt du blocage, que nous appelons de nos voeux. En l'absence d'une telle décision, là encore- Mme la Première ministre l'a annoncé -, l'État prendra ses responsabilités et décidera des réquisitions nécessaires pour que chacun puisse retrouver un quotidien

En réalité, nous sommes face à un dilemme : une troisième étoile sur le maillot bleu vaut-elle toutes les compromissions ? Car, des compromissions, il y en a eu et il y en a encore. En 2010, Kylian Mbappé n'avait que 12 ans, mais, à cette époque, Nicolas Sarkozy oeuvrait déjà avec succès pour que la monarchie qatarie se voie attribuer l'organisation de l'événement. Douze ans plus tard, on s'apprête à jouer la plus grande compétition de football sur les cadavres de 6 500 travailleurs qui ont participé à la construction de stades climatisés. Douze ans plus tard, les droits humains n'ont pas progressé au Qatar, les minorités sexuelles sont toujours persécutées, les femmes ne sont pas libres et l'esclavage continue. ans plus tard, le climat prend la trajectoire d'un chaos global et on continue d'organiser de grands événements sportifs dans le déni climatique, en dépit de toutes les alertes, de toutes les catastrophes, de tous les emballements, de tous les drames qui surviennent. sans doute, madame la ministre, que vous n'êtes pas comptable des compromissions passées, mais la France s'apprête à exporter, demain, son savoir-faire en matière de sécurité, en mettant au service de la dictature qatarie 220 gendarmes et agents de la sécurité civile, tous des hommes, bien entendu, pour ne pas choquer le rigorisme religieux des émirs Pourtant, au-delà du rayonnement de nos équipes nationales, le sport français devrait être un réel vecteur d'engagement en faveur des droits humains et du climat. Ma question est donc la même que celle que je posais à votre prédécesseur voilà quelques mois, à l'occasion des jeux Olympiques au pays du génocide ouïghour si nos joueurs n'ont pas à assumer les choix politiques de la France, allez-vous, de votre côté, au moins boycotter diplomatiquement cette Coupe du monde de la honte et de la compromission ? Allez-vous enfin engager votre ministère dans une réelle diplomatie sportive au service du climat et des droits humains ?

dans un tout autre contexte. Aujourd'hui, l'urgence écologique est, bien entendu, plus prégnante que jamais et nous souhaitons que le Qatar fasse tout ce qu'il doit faire pour tenir l'objectif de neutralité carbone qu'il a affiché pour ce Mondial.

nous avons pris l'engagement de faire de nos jeux Olympiques et Paralympiques les jeux les plus écologiques de l'histoire. Nous tiendrons cet engagement, de la même façon que, dans la foulée du plan de sobriété énergétique porté par la ... Vous avez ! La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. et Territoires. Monsieur le ministre de la santé, une autre pénurie menace la France : celle des médicaments. L'alerte lancée récemment à ce sujet par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé concerne les traitements les plus courants du diabète de type 2, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Depuis janvier dernier, les ruptures d'approvisionnement des officines augmentent de manière constante et sont en passe d'être multipliées par deux. Au-delà des antidiabétiques, les médicaments de lutte contre l'hypertension ou anticancéreux sont également concernés par ces tensions, mais cela touche de plus en plus de médicaments. De manière plus générale, ce sont les princeps ou les médicaments qui n'ont pas de solution thérapeutique de substitution qui connaissent ces difficultés. Les témoignages émanant du terrain sont clairs : il manque de plus en plus de molécules chez les pharmaciens. En 2018, déjà, notre collègue Jean-Pierre Decool avait soulevé ce problème à l'occasion d'une mission d'information demandée par le groupe Les Indépendants. Des pistes d'amélioration de notre système avaient été proposées. Les causes de ces pénuries sont multiples et l'aggravation de la situation est due, en partie, aux fortes tensions déclenchées par la pandémie de covid-19 et, plus récemment, par la guerre en Ukraine. Beaucoup de nos médicaments proviennent d'Asie. Les matières premières pour les fabriquer sont quasiment toutes hors de l'Union européenne. Nos chaînes de distribution ne sont pas assez efficaces. C'est un problème de souveraineté pour la France et pour l'Europe ; nous devons produire nos médicaments. Les ruptures de stock et les tensions sur les approvisionnements nous fragilisent. Nous risquons des drames humains. Nous ne pouvons pas l'accepter. Monsieur le ministre, quelles réponses conjoncturelles et surtout structurelles comptez-vous apporter pour lutter contre ces pénuries ? L'échelon européen n'est-il pas incontournable ? bonne question ! La parole est à M. le ministre de la santé et de la prévention. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Mélot, le médicament est un secteur stratégique, essentiel pour notre pays, qui répond à plusieurs enjeux

nous nous trouvons désormais, il est devenu préférable, pour nombre d'entreprises, de cesser de produire, voire de fermer ses portes, plutôt que de continuer de créer de la richesse, car produire fait perdre de l'argent

sans énergie, donc sans activité, au 1 janvier prochain. En effet, sur le marché, les contrats à terme sont devenus inexistants. Les offres, quand elles existent, ne sont valables que quelques heures et ne sont pas économiquement accessibles. Le marché, sans repères, est devenu imprévisible et personne- personne ! -ne semble vouloir saisir la bride de ce cheval devenu fou ... Les chefs d'entreprise sont seuls. L'un d'eux m'a écrit hier : « Mais qu'attendent-ils ? Nous mourons et nous mourons de mort subite

... Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour apporter une solution simple, massive et extrêmement rapide en soutien de nos entreprises ?

est menacée. Quelles mesures allez-vous prendre ou avez-vous déjà prises pour soutenir les agriculteurs dans cette période extrêmement difficile ? La parole est à M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur

depuis un certain temps, nos compatriotes regardent avec effarement tourner le compteur des pompes à essence. Et dans le même temps, les actionnaires regardent grimper les chiffres des dividendes avec ravissement. Les prix des carburants s'emballent, la spéculation sévit et TotalEnergies s'enrichit, y compris grâce à l'argent public du bouclier tarifaire. L'entreprise a enregistré plus de 10 milliards d'euros de bénéfice net au premier semestre de cette année, ce qui valut aux actionnaires, le 28 septembre dernier, de bénéficier d'un dividende exceptionnel de 2,6 milliards d'euros. TotalEnergies deviendra demain TotalBénéfices ! Les salariés des groupes pétroliers demandent légitimement leur part de cette « réussite » et revendiquent une hausse de leurs salaires.

Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps de faire pression sur les directions des groupes TotalEnergies et ExxonMobil. À l'évidence, leur demander aimablement « un geste de bonne volonté » ne suffit pas. Cela est d'autant plus nécessaire que, face aux salariés, le Gouvernement brandit la menace inacceptable de la réquisition.

de par votre appartenance politique, de par les combats que vous avez menés, je vous sais plus attaché que quiconque ici ... À la CGT ! ... à la qualité du dialogue social et au respect des accords obtenus à travers ce même dialogue social. Monsieur le sénateur, je vous invite à considérer une situation

pour la réplique. Les salariés des groupes concernés ne demandent pas une hausse de 52 % de leurs revenus, à l'image de celle que le PDG de TotalEnergies s'est octroyée. Ils demandent leur part légitime. En cette rentrée de forte inflation, la question du pouvoir d'achat est devenue la première préoccupation de nos concitoyens. Comment pourrait-on s'étonner de leurs revendications ? Vous allez déposer deux amendements au projet de loi de finances visant à dégager, nous dit-on, 200 millions d'euros : c'est très, très loin du compte. Il faut taxer fortement les superprofits pour aider les salariés, les retraités, les entreprises et les collectivités.

en réponse à ma demande de juillet dernier. Je voudrais aussi profiter de cette période de consultations générales pour attirer votre attention sur la situation sanitaire à Wallis-et-Futuna. Comme vous le savez, monsieur le ministre, depuis 2005, aucune politique de prévention n'a été mise en place par l'Agence de santé, ce qui a permis à des maladies telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires de se développer sur le terrain. sociales (Igas) de 2019 avait pourtant préconisé de mettre l'accent sur la prévention. Mais ce rapport est resté très officieux, et ce au détriment de notre population. Je souhaite ici m'assurer que la conférence de santé se tiendra au premier semestre 2023 à Wallis-et-Futuna et qu'elle associera toutes les instances locales et l'ensemble de la population. ailleurs, monsieur le ministre, le lancement du volet santé du Conseil national de la refondation (CNR-santé) doit aussi être l'occasion de restaurer le lien de confiance rompu entre la population et l'Agence de santé. Nos sensibilités locales ne sont pas entendues ; les professionnels de santé fuient le territoire. Je souhaite enfin attirer votre attention sur deux autres situations prioritaires. Premièrement, celle des dialysés, qui ont besoin du renouvellement des huit générateurs d'hémodialyse devenus obsolètes et d'un véhicule adapté pour leur transport.

comment le Gouvernement entend-il aider Wallis-et-Futuna à se doter d'un système de santé et d'une organisation des soins adaptée aux besoins de la population ? La parole

En tant que ministre de la santé et de la prévention, mais aussi en tant que médecin, je ne peux accepter une situation où le manque de prévention ne permet pas de répondre aux besoins de santé de la population

chute des surfaces de blé, recul du cheptel laitier faute d'un revenu suffisant pour les éleveurs ... C'est incontestable, la ferme France produit de moins en moins. Depuis 2017, vous prônez la montée en gamme

Vous mettez en danger notre souveraineté alimentaire en condamnant certains de nos concitoyens à n'acheter que des produits importés. On marche sur la tête ! Notre manque de compétitivité est à la racine de nos maux coût de la main-d'oeuvre, surtransposition, suradministration, manque d'investissements, signature d'accords de libre-échange qui condamnent nos agriculteurs

à ne manger qu'un jour par semaine ! Plutôt que la décroissance, il nous faut un vrai choc de compétitivité ! Madame la Première ministre, après le théâtre Guignol du col roulé et de la doudoune, enfilez enfin vos bottes pour comprendre la situation préoccupante de notre agriculture. La parole

et Républicain. Monsieur le ministre de l'intérieur, la commission des lois du Sénat a décidé la création d'une mission d'information pour examiner l'opportunité de la réorganisation de la police judiciaire On aurait pu imaginer que cette initiative, qui a inspiré l'Assemblée nationale, vous permette de recréer les conditions d'un dialogue serein. Que constate-t-on un mois après ? La mobilisation de la PJ, que le directeur général de Fâché par une vidéo, ce dernier a d'ailleurs limogé le patron de la PJ marseillaise. Résultat : la contestation s'étend et devient visible dans la rue. Vous citez des rapports parlementaires et des ministres pour justifier votre réforme. Mais aucun de ces rapports ni aucun de vos prédécesseurs n'était parvenu à inquiéter l'ensemble de la PJ. Même la PJ parisienne, dont vous rappelez qu'elle n'est pas concernée, soutient le mouvement. Vous incriminez la proximité des élections syndicales pour justifier ce climat, tout en affirmant que l'ensemble des syndicats soutient votre réforme ... Hier, même les très discrets procureurs généraux ont renouvelé leur opposition à cette réforme, considérant que ce projet constitue une « remise en cause de la place accordée à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle dans un État de droit ». Monsieur le ministre, n'est-ce pas le moment de revoir votre copie ?

Le fait de nommer [ ...] des directeurs départementaux de la police nationale a été accueilli avec curiosité, parfois avec inquiétude, y compris chez certains fonctionnaires de la police nationale, notamment les commissaires.

Aujourd'hui, les services de la police judiciaire sont placés sous l'autorité des chefs de service régionaux de police judiciaire et du directeur central de la police judiciaire. Le préfet, en tant que chef de l'ensemble des services de l'État et parfois des services du ministère de l'intérieur dans le département, aura autorité sur eux, dans l'exacte mesure où il peut avoir autorité sur des services de fonctionnaires,

Monsieur le ministre, vous me renvoyez à ce qui s'est passé voilà trente ans ; je vous parle d'aujourd'hui. Notre mission sénatoriale se prononcera au fond, mais,, il y a un problème de méthode. Les policiers ne réagissent pas par corporatisme. Ce qui est en jeu, c'est la séparation des pouvoirs et le modèle français d'enquête. la police judiciaire sous l'autorité du préfet, c'est courir le risque d'abandonner les enquêtes complexes, la lutte contre la criminalité organisée, devant le flux inexorable du quotidien. Monsieur Darmanin, nous connaissons votre grand talent. Mais aujourd'hui, à part vous, personne ne semble soutenir cette réforme.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le 13 juillet dernier, je vous interrogeais en commission de la culture sur mes vives inquiétudes concernant votre ministère et la situation de l'école en France après votre nomination. Je vous demandais de nous rassurer ; trois mois plus tard, mes inquiétudes demeurent. Le Président de la République a décidé de lancer lui-même l'année scolaire en réunissant les recteurs d'académie. Pensez-vous que l'élan pour transformer l'école doit être si puissant qu'il ne puisse venir que du chef de l'État ? Cette verticalité interroge sur votre rôle et vos marges de manoeuvre, tout en posant de nouveau la question : rupture ou continuité après votre prédécesseur ? Monsieur le ministre, les faits et les réalités vous rattrapent. La rentrée scolaire n'a pas été à la hauteur : il n'y avait pas un enseignant devant chaque classe et d'aucuns étaient même formés en quatre jours. Les difficultés de terrain se multiplient : désenchantement général des enseignants et hausse des signalements pour atteintes à la laïcité. Votre communication prudente est, là encore, insuffisante. La communauté éducative a besoin de directives claires, d'une volonté politique ferme Vos récents propos tenus à l'étranger m'ont également inquiété. Monsieur le ministre, vous avez pensé pouvoir affirmer à New York qu'il y avait des traces d'anti-américanisme dans le discours politique français. Vous avez suggéré l'impossibilité d'évoquer avec nuances les inégalités raciales dans notre pays. Non, monsieur le ministre, la France n'est pas raciste. Nous sommes, nous aussi, sensibles aux questions d'inégalités. N'abîmez pas à l'étranger nos principes fondateurs. Cessez de vous positionner comme universitaire militant, ne tentez pas de nous imposer un « wokisme de salon », cher à notre président Retailleau, incompatible avec vos responsabilités politiques. Soyez ministre enfin les seules questions qui s'imposent : quelle est votre vision de l'école ? Où voulez-vous emmener les enseignants et nos enfants ?

Je suis aussi de ceux qui estiment que la lutte contre les différentes formes de discrimination, contre le racisme, contre l'antisémitisme et la haine anti-LGBT n'affaiblit pas la République, mais la renforce. C'est une manière d'exprimer

J'ai aussi dit mon attachement à une République fidèle à ses valeurs, celles des droits humains, et qui, non contente d'inscrire ses principes au frontispice de ses bâtiments, les met en oeuvre. En tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, je ne suis pas simplement attaché à la lettre, mais aussi à la mise en oeuvre concrète des politiques de cohésion sociale, de réussite pour tous les élèves et d'égalité des chances. Des actes ! Monsieur Monsieur le sénateur, ne voyez ici point de « wokisme de salon », mais mon seul attachement, en tant que citoyen, en tant que ministre, aux valeurs universelles de la République.

de la République. Vos mots ne répondent ni à l'effondrement des connaissances et à la crise de la transmission ni aux immenses défis posés à l'école. Monsieur le ministre, apportez à votre ministère, apportez aux Français la sérénité dont nous avons tous

Madame la ministre, nombreux sont les maires confrontés au fléau des déserts médicaux. Or la transformation du en n'est pas près de produire ses effets. Face à cette situation, les maires cherchent désespérément des médecins français ou européens pour leurs administrés. Mais devant les échecs à répétition, ils se mettent finalement en quête de médecins hors Union européenne, quand ils ne sont pas sollicités par ces mêmes médecins. Ceux d'entre eux qui ont des pistes pour faire venir un médecin étranger francophone abandonnent souvent leurs démarches, lassés des difficultés administratives. C'est à se demander si tout n'est pas fait pour décourager la venue de ces médecins en asphyxiant les maires par des démarches complexes, dont ils n'arrivent souvent pas à voir l'issue. Pour ne pas paraître autocentré sur mon département, bien qu'il soit tout autant concerné, je vais prendre l'exemple de la commune de Latour-de-France, dans les Pyrénées-Orientales- mes collègues Jean Sol et François Calvet connaissent très certainement cette histoire. Cette ville n'a plus de médecin généraliste depuis le 22 octobre 2021, situation devenue malheureusement banale dans nos territoires ruraux. Le maire a réussi à trouver un médecin pour sa commune, mais celui-ci est Libanais et exerce actuellement à Beyrouth.

Cet exemple n'est, hélas, pas isolé et c'est bien l'ensemble de nos territoires ruraux qui sont confrontés à ces difficultés. Compte tenu de la tension qui règne en France en matière d'accès aux soins, ne devrions-nous pas songer à favoriser l'implantation de ces médecins non communautaires, en facilitant, de façon dérogatoire, les procédures administratives ? Cela permettrait d'apporter une réponse, même partielle, à la crise des déserts médicaux. Pourquoi, par exemple, ne pas organiser cinq à dix concours d'évaluation des connaissances et compétences par an, au lieu de un à deux actuellement ? Répondre à la pénurie de médecins passera forcément par de multiples dispositifs. Celui-ci en est un parmi tant d'autres. Aussi, madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer ce que compte faire le Gouvernement en la matière ? La parole

La crise sanitaire a malheureusement empêché l'organisation des commissions d'autorisation en raison de la forte mobilisation des membres des jurys, qui sont des professionnels de santé, et des candidats eux-mêmes, dans les établissements de santé,

afin de traiter le plus grand nombre de dossiers avant la date butoir du 31 décembre 2022 posée dans la loi OTSS. Malheureusement, nous savons que ces 2 400 dossiers ne pourront être traités, raison pour laquelle le Gouvernement a déposé,

défiance populaire envers la parole publique atteint des sommets, mieux vaut une République exemplaire. Permettez-moi donc de m'interroger sur une contradiction de votre gouvernance : une règle, certes informelle, mais inlassablement répétée depuis vingt-cinq ans, veut qu'un ministre

Y aurait-il donc des ministres privilégiés, de fortes têtes capricieuses, un problème d'autorité de votre part ? Madame la Première ministre, comptez-vous enfin faire appliquer la

Les braconniers étant les meilleurs gardes-chasses, Mme la Première ministre m'a demandé de répondre à votre question, monsieur le sénateur. Tout d'abord, je veux vous dire, au nom du Gouvernement et de Mme la Première ministre, que les règles seront respectées. Plusieurs ministres ont déjà

L'exemplarité ne se proclame pas, elle se pratique et Républicain. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Face à l'internationalisation du conflit en Ukraine et à sa dramatique densification, quelles sont les initiatives, les actions, que compte mener la France ? Allons-nous continuer à rechercher une issue diplomatique ? Allons-nous décider d'augmenter notre contribution humanitaire, financière ou militaire ? Cela en prend le chemin, puisque la France vient d'annoncer qu'elle renforçait sa présence militaire en Roumanie dans le cadre de l'Otan. Allons-nous tenter de peser sur le G7 ? Mais que peut décider le G7, réuni en urgence, sinon réitérer un affichage de solidarité ? Allons-nous faire la promotion de nouvelles sanctions ? Je partage les mots du Président de la République : nous assistons à un changement profond de la nature de cette guerre, la mesure où le Bélarus s'apprête à véritablement devenir la base armée et le fer de lance de la politique russe dans la gradation du conflit. Ils seraient bien avisés de ne pas entrer dans la guerre. » Ce sont vos propres mots, madame la ministre. Minsk, ce n'est pas seulement le nom d'accords qui n'ont pas abouti, c'est surtout la capitale d'un pays martyr, dans l'angle mort de nos actualités, alors que s'y joue la vie de plusieurs centaines de prisonniers politiques, dont je veux faire résonner le nom et saluer le courage. Madame la ministre, à l'aune d'un conflit qui nous concerne tous, à l'échelle internationale, comment comment apprécier le fléchissement de la politique du Bélarus ? La parole Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Muriel Jourda, vous avez raison, depuis lundi, la Russie a lancé une série de frappes sur le territoire ukrainien, qui visent principalement les infrastructures civiles et qui ont sans doute pour objectif d'atteindre le moral de la population ukrainienne. La France l'a réaffirmé, son soutien à l'Ukraine se poursuivra et s'intensifiera.

mais aussi politique et diplomatique, car il y a un agresseur et un agressé. Hier, les dirigeants du G7 ont condamné les dernières attaques russes, qu'ils ont qualifiées de crimes de guerre. Ils ont déclaré que leurs responsables devront rendre des comptes. Ce soir même ou dans la nuit, l'Assemblée générale des Nations unies se prononcera sans ambiguïté sur l'annexion illégale du territoire ukrainien par la Russie, ce qui montrera une fois de plus l'isolement l'isolement de cette dernière. J'ai répondu indirectement, madame la sénatrice, à votre question sur le Bélarus, lequel, en effet, ne doit pas s'engager davantage dans son soutien à l'opération illégale menée par la Russie. En outre, je le rappelle, l'Union européenne a mobilisé déjà plus de 9 milliards d'euros. Elle a porté la Facilité européenne pour la paix à 2,5 milliards d'euros et a adopté huit séries de sanctions, pour peser sur l'effort de guerre russe. Je vous le dis, il y aura,

Vial, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école est une priorité. C'est aussi un défi pour lequel nous sommes tous mobilisés depuis la loi de 2005. Pourtant, cette rentrée scolaire ne s'est pas déroulée, pour beaucoup de ces enfants, comme toutes les autres. En effet, depuis septembre, à la suite d'une décision de justice sollicitée et obtenue par votre prédécesseur, l'État s'est désengagé du suivi et de la prise en charge de ces enfants à besoins particuliers sur le temps périscolaire et celui de la cantine. S'il s'agit, une fois encore, d'un transfert de charges de l'État vers les collectivités, sans compensation, la question financière n'est pas, de très loin, le problème principal. Le plus important est le transfert de responsabilité

Monsieur le ministre, probablement faudra-t-il revoir en profondeur la politique d'inclusion des enfants et adolescents en situation de handicap, dont le nombre a plus que quadruplé en vingt ans, pour atteindre 430 000 enfants à cette rentrée, soit environ 3,5 % des effectifs totaux, soit un élève en moyenne par classe Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à vous engager à mettre en place des conventions de mise à disposition d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps de midi, signées entre votre ministère et les maires, ce qui favoriserait leur recrutement et leur formation et permettrait un suivi de qualité des enfants concernés ? Le Conseil d'État recommande cette solution, la loi la permet, les maires de France la réclament, Jean-Michel Blanquer l'avait promise ! Pourtant, votre administration refuse de la mettre en place De fait, depuis la rentrée, des enfants ne sont pas accompagnés, les familles sont inquiètes, les équipes éducatives sont déstabilisées. Monsieur le ministre, le plus grand handicap, c'est d'être absents là où notre présence est utile.

vous avez raison, l'école inclusive est l'une des grandes réussites du système scolaire, avec l'inclusion de plus de 430 000 élèves en situation de handicap

survenir très tard, jusqu'à la dernière minute avant la rentrée. Nous devons donc en quelque sorte courir derrière une marée de notifications, ce qui crée des difficultés pour les familles et les élèves, je le reconnais volontiers. Vous faites allusion à une question particulière, qui est celle de la pause méridienne. Vous avez eu raison de mentionner l'arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 2020, qui nous enjoint de rémunérer les AESH sur le temps scolaire et non pas sur le temps périscolaire.

évidemment l'intérêt qu'il y a à maintenir la continuité, particulièrement pour certains types de handicaps. Je pense ici aux enfants en situation autistique, qui représentent

Leur doléance est simple : ils réclament des embauches parce que notre système est totalement obsolète. Il faut encore des personnes physiques pour assurer l'aiguillage des trains. Sur ce sujet de modernisation du rail, nous avons quarante ans de retard. Moderniser notre rail, c'est mettre en place de nouveaux systèmes de signalisation, à commencer par le Système européen de gestion du trafic ferroviaire. C'est aussi regrouper la gestion des 2 200 aiguillages dans seize postes de commande centralisés du réseau digitalisé. C'est enfin numériser le système de gestion de transport. Pour combler cette lacune, un énorme effort d'investissement doit être consenti aujourd'hui. Aujourd'hui correspond au pire moment, puisque la flambée du coût de l'électricité plombe les dépenses de fonctionnement des autorités organisatrices de transports. À titre d'exemple, en Île-de-France, ce surcoût représente 950 millions d'euros pour boucler le budget de 2023. L'essentiel de cette somme n'étant pas financé, le spectre récemment agité d'un passe Navigo augmenté à 100 euros inquiète. Je le dis ici, car je sais que nous partageons tous ce point de vue, il n'est évidemment pas question de pénaliser davantage les usagers. Dans ces conditions, il est légitime de craindre un effet de vases communicants entre les choix d'investissement et de fonctionnement, ces derniers phagocytant les premiers. Ce faisant, il s'agit également d'une remise en cause de notre chemin vers la neutralité carbone, car le report modal sur le train est un axe clé de la stratégie gouvernementale. Aussi, monsieur le ministre, avez-vous identifié une telle menace et comment comptez-vous y répondre d'un point de vue budgétaire ?

cas, par les coûts de l'énergie. Parce que le sujet est grave et important, nous devons être très clairs vis-à-vis de nos concitoyens sur les responsabilités, pour ne pas être dans un jeu de postures. Qui est responsable de l'organisation des transports dans la région Île-de-France, comme dans les autres régions ? C'est Île-de-France mobilité, c'est-à-dire la région elle-même.

La présence de la police municipale ne doit pas être prétexte pour l'État à se désengager de ses missions régaliennes, y compris la police de proximité. Toutefois, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante peut autoriser le maire à signer avec l'État, pour une durée n'excédant pas celle du mandat de cette assemblée, une convention de partenariat entre la police municipale et la police nationale.

aussi nous assurer de la réalité de cette intention. En effet, en lisant entre les lignes, on s'aperçoit que cette politique d'ouverture est souvent mise au service d'une autre politique, celle du résultat, la première étant censée donner à la seconde une justification académique. Or cela ne peut ni ne doit être la base d'une relation saine et constructive entre ces deux mondes. Nous rappelons ainsi que le monde de la recherche ne saurait être

en leur fournissant tous les documents nécessaires à la réalisation de leurs travaux. Nous considérons aussi que cette ouverture doit se faire jusqu'au coeur des institutions. C'est pourquoi nous vous proposons qu'au sein de la future académie de police prévue dans le rapport des heures de cours soient dispensées aux policiers en formation par des chercheurs en sociologie ou en toute autre branche des sciences humaines et sociales ayant rapport avec les questions de sécurité. L'ouverture au monde de la recherche est salutaire, mais les conditions dans lesquelles celle-ci s'opère doivent être précisées. Quel est l'avis de

et rappeler le principe de la liberté de la recherche, c'est, sinon superfétatoire, du moins superflu ! Le rapport annexé n'a pas vocation à aller à l'encontre des grands principes qui régissent la recherche et la politique de l'État est déjà une politique d'ouverture des données, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de données sensibles. Avis défavorable.

nous ouvrons le ministère de l'intérieur au monde de la recherche, et c'est une excellente chose. Ce n'est pas nous qui allons sélectionner les chercheurs ; mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas vous non plus ... Avis défavorable.

ou de textes plus récents. Peu importent les rappels du Conseil constitutionnel quant au nécessaire encadrement des technologies intrusives : le Gouvernement ne manque pas de revenir à la charge de manière purement dogmatique.

massive de la population. Là encore, nous sommes bien conscients de l'absence de portée normative du rapport. Mais il s'agit bien d'un rapport d'orientation, et notre groupe trouve plus que nécessaire d'y inscrire cette interdiction. Les débats cette interdiction. Les débats suscités par cette technologie ne font que grandir : en janvier 2020, dans la prépublication de son livre blanc sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne envisageait la mise en place d'une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs. Le présent amendement est directement inspiré des travaux de notre collègue députée Paula Forteza et du groupe écologiste de l'Assemblée nationale, qui souhaitaient un moratoire sur l'usage de la reconnaissance faciale à des fins d'identification des individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu'à ce que des garanties suffisantes soient établies en matière de sécurité et de libertés fondamentales. Les données faciales sont des données biométriques sensibles et constituent des informations irrévocables, à l'inverse de nos mots de passe ou adresses mail. Elles sont par définition uniques et inchangeables en cas de vol ou de compromission. Une protection accrue de ces données doit être mise en place, notamment quant aux personnes ayant accès à ces données. Cela soulève donc des enjeux cruciaux en matière de libertés publiques, d'éthique et de consentement. Les interrogations, les doutes et les peurs découlent en partie de la non-maîtrise de cette technologie et de certains usages débridés de la part d'entités privées et publiques. D'une part, la reconnaissance faciale n'est pas à ce jour une technologie totalement mûre et possède encore de nombreux défauts techniques ; il existe notamment des biais lorsqu'il s'agit de minorités ethniques, de femmes et de jeunes. D'autre part, cette technologie peut engendrer des dérives mettant en danger nos libertés et notre démocratie, comme le démontrent les cas de la répression des manifestations à Hong Kong ou de la surveillance de la minorité ouïghoure par la Chine. Le déploiement d'un système général de reconnaissance faciale pourrait mettre fin à toute possibilité d'anonymat, ce qui irait à l'encontre de notre conception des libertés de circulation et d'expression. Je redis les choses : la reconnaissance faciale est actuellement interdite en France. M. le ministre s'est exprimé hier sur le sujet sans aucune ambiguïté.

les lignes rouges qu'il faut tracer en la matière et les conditions dans lesquelles certains algorithmes pourraient être utilisés une loi d'expérimentation, des mesures de transparence et le contrôle d'une autorité indépendante.

les attentes de l'ensemble de la société civile en matière de numérique, nouer une relation de confiance avec les forces de sécurité, coconstruire un cadre normatif approprié et mener une analyse d'impact rigoureuse de la reconnaissance faciale. J'ajoute, à l'attention de notre rapporteur,

Monsieur Durain,

Va-t-on continuer longtemps à s'interroger : faut-il ? ne faut-il pas ? Je partage avec les membres de mon groupe quelques convictions simples : les nouvelles technologies sont là et bien là, et ce souvent contre nous.

Un usage proportionné de ces outils est donc nécessaire, et il est temps que la loi dise ce qui est possible, ce qui est souhaitable, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas- et nous arrêterons de débattre dans le vide.

Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur les régions et territoires d'outre-mer, la Guyane a le triste privilège d'avoir à en affronter qui lui sont spécifiques, comme l'orpaillage illégal et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). C'est une véritable atteinte à la souveraineté de notre pays que commettent les brésiliens et les pêcheurs surinamais, guyaniens ou brésiliens : ils profitent de l'immensité du territoire et de la faible présence des forces de sécurité pour venir piller ces ressources. En outre, par la pollution que causent les orpailleurs clandestins et par l'épuisement des écosystèmes sous-marins que provoquent les bateaux de pêche INN, cette criminalité porte une atteinte grave à l'environnement qui, à terme, pourrait être irréversible. Enfin, les filières d'approvisionnement des sites d'orpaillage clandestin font appel à des réseaux criminels qui volent et parfois violentent la population guyanaise. Quant aux pêcheurs illégaux, ils n'hésitent plus à s'attaquer en pleine mer aux pêcheurs guyanais et à leur voler leur matériel, voire leur pêche. C'est toute la filière économique guyanaise de la pêche qui s'en trouve fragilisée. Dès lors, il semble indispensable que la lutte contre ces deux fléaux fasse partie des priorités des autorités en matière de lutte contre la criminalité pour les prochaines années.

pas plus qu'une procédure numérique, ne saurait satisfaire nos concitoyens victimes ni les personnes ayant commis un délit. En effet, les assistants d'enquête seront des profanes en matière de procédure pénale et de gestion des prévenus dans un commissariat, ce qui risque fortement

ne sera pas traitée par un algorithme décidant ou non du classement sans suite. Cette création d'assistants d'enquête vise en réalité, selon nous, à pallier un déficit de formation ; en la matière, nous proposons, quant à nous, un triplement du budget.

L'ancienne adjointe du Défenseur des droits en charge de la déontologie, Mme Claudine Angeli-Troccaz, a expliqué la dangerosité d'une telle arme et les risques disproportionnés qu'elle fait courir dans le contexte des manifestations Dans une foule mouvante, cette arme imprécise n'atteint généralement pas sa cible et occasionne des blessures graves. Les utilisateurs disent eux-mêmes qu'elle est difficile à maîtriser et que sa marge d'incertitude est grande. Le ministère de l'intérieur a toujours été frileux quant à l'encadrement de cette technique, n'émettant le 23 janvier 2019 que des préconisations molles visant à doter « dans la mesure du possible » les tireurs équipés de LBD « d'une caméra-piéton à fixation ventrale de préférence Le maintien de l'ordre doit s'inspirer de doctrines moins frontales. Si le schéma du maintien de l'ordre présenté en décembre 2021 l'évoque, la place réservée aux armes de force intermédiaire reste trop importante. En effet, au cours de l'année 2019, lors des manifestations des « gilets jaunes », de nombreuses personnes ont été mutilées par ces deux armes.

mutilations. Au regard des objectifs du maintien de l'ordre, l'usage de ces armes au cours de manifestations s'avère donc totalement disproportionné. Face à la multiplication des incidents, le présent amendement, inspiré des travaux de différents groupes parlementaires, vise à supprimer l'utilisation de telles armes lors d'opérations de maintien de l'ordre.

Il n'est ni supportable ni acceptable que les forces de l'ordre fassent régulièrement la « une » des journaux nationaux, et désormais internationaux, du fait de la répression violente et inadaptée d'événements en tous genres. Qu'il s'agisse d'un afflux de supporters anglais pacifiques au Stade de France, des rassemblements de « gilets jaunes », des manifestations- voire des rassemblements -en soutien aux femmes iraniennes, la doctrine est toujours la même et tient en quelques mots : lacrymogènes, grenades de désencerclement, matraques et nasses. Ces méthodes, inefficaces, ont atteint leur limite. Il est devenu très compliqué de manifester dans ce pays. La doctrine de maintien de l'ordre, qui consiste à considérer les manifestants comme des éléments hostiles, d'où qu'ils viennent, n'aboutit qu'à une montée en tension et au désordre. L'expérience du Stade de France a été éclairante sur l'inefficacité de cette doctrine. Il est temps d'en finir avec cette militarisation à outrance du maintien de l'ordre et de concevoir des stratégies de désescalade et de dialogue. Si de tels événements se sont produits au Stade de France, que se passera-t-il lors des jeux Olympiques de 2024, quand le monde aura le regard braqué sur nous ? Il est urgent de changer la doctrine non seulement pour la sécurité des manifestants et des participants aux rassemblements, mais aussi pour les policiers et gendarmes qui subissent cette montée en tension permanente. Quel

dont ne dispose pas un agent de police judiciaire (APJ). C'est notamment lui qui prend la décision de recourir à une mesure de garde à vue, sous l'autorité du ministère public, et qui se transporte au domicile du mis en cause en cas de flagrance. De telles décisions nécessitent mesure et maturité. Il n'est donc en aucun cas judicieux d'abaisser les seuils d'exigence et de trop faciliter l'accès à cette profession de très grande responsabilité. Quel

examinons sous forme d'amendements, dans le cadre d'une procédure législative, les dispositions générales d'un rapport qui n'a pas de caractère législatif. Il me semble donc qu'il y a eu une erreur de manoeuvre de la commission, laquelle a consenti à ce que tout cela donne lieu à une

M. Fabien Gay. Puisque j'ai eu une mauvaise note, j'y retourne ... Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section intitulée « Alléger le formalisme procédural et simplifier la procédure pénale ». Vous le savez, nous rejetons formellement l'allégement du formalisme procédural et la simplification de la procédure pénale, laquelle doit préserver un équilibre entre l'objectif de recherche, la poursuite des infractions, et la garantie de la liberté et des droits des citoyennes et des citoyens. Nous refusons la dématérialisation du dépôt de plainte et de son suivi. La volonté d'aller vite s'entend, que ce soit pour les victimes ou pour les enquêteurs. Mais encore faut-il ne pas priver les victimes d'un accueil humain et physique Et quand bien même l'utilisation d'une telle dématérialisation servirait uniquement pour les atteintes aux biens, l'aspect cathartique pour la victime du déplacement au commissariat n'est, selon nous, pas à négliger. L'amendement n° 226, présenté

Selon le professeur de droit Olivier Cahn, « le recours à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle transfère aux forces de l'ordre non seulement la charge de la qualification de l'infraction mais l'opportunité de décider d'une répression minorée et accélérée, ce qui privera le parquet de la possibilité d'exercer son pouvoir d'opportunité des poursuites La généralisation de l'amende forfaitaire délictuelle va étendre l'application de mesures intrusives ou coercitives, prises sans contrôle préalable d'une autorité juridictionnelle, au mépris des dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale, lequel prévoit qu'il revient au procureur d'apprécier l'opportunité des poursuites.

Le Syndicat des avocats de France (SAF), de son côté, pointe un autre élément. Il se dit très inquiet quant aux difficultés de faire un recours contre ces amendes. Le recours n'est pas suspensif, et l'on ne prévient pas les intéressés qu'ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police.

Par cette généralisation, nous assistons à une politique de contournement de la justice répressive, dont les potentielles dérives ne feront qu'accroître le sentiment de défiance des citoyens vis-à-vis de leur police. Or c'est un point que nous voulions mettre en avant lors de cette discussion.

Assassi. Nous considérons que l'idée d'introduire des délégués du procureur dans les commissariats et les gendarmeries est bonne, car cette mesure contribue à l'efficacité de l'enquête. Pour autant, elle n'est pas satisfaisante. Pour renforcer les droits des gardés à vue, mais également des victimes, il convient d'introduire au sein des commissariats et des gendarmeries des agents de police judiciaire ne prenant pas part à l'enquête, et dont la mission serait de vérifier le respect des garanties procédurales tout au long de la garde à vue. Nous considérons, à vue. Nous considérons, en outre, qu'il est nécessaire d'aller dans le sens d'un renforcement de la procédure pénale et non d'une simplification. Les métiers de la sécurité intérieure doivent pouvoir être exercés sereinement c'est pourquoi l'instauration d'un agent de police judiciaire extérieur à l'enquête permettrait de prévenir tout vice de procédure et consoliderait celle-ci, en évinçant les causes de nullité susceptibles de l'entacher. Ainsi, les agents de police judiciaire exerceraient leurs fonctions sans cette épée de Damoclès : voir une procédure annulée pour ne pas avoir respecté certaines obligations procédurales.

tend donc à développer les mesures que les forces de l'ordre pourraient mettre en oeuvre afin d'être formées sur les conséquences réelles du changement climatique, mais aussi afin de prévenir, contrôler et sanctionner les atteintes à l'environnement à une plus grande échelle, et de consacrer ainsi le rôle de protecteur de la nature de la police. Celle-ci a un réel rôle à jouer dans ce domaine : sensibiliser à la protection de notre environnement ; protéger notre propriété commune ; contrôler et sanctionner ceux et celles qui polluent en toute impunité. Ces mesures seront très utiles aux collectivités territoriales et à tous nos territoires.

de sensibilisation, avec la participation de la population- on parle de risques industriels, évidemment. Cette politique doit être saluée, notamment lorsqu'elle témoigne, comme c'est le cas dans le rapport, d'une prise en compte des conséquences du dérèglement climatique qui touche déjà, et touchera encore plus fortement à l'avenir, Cette prise de conscience salutaire des enjeux de résilience peut être encore améliorée si on lui adjoint un autre risque, dont on parle peu, mais qui, pourtant, est loin d'être nul au vu de la politique énergétique de notre pays : le risque nucléaire et radiologique. Qu'ils soient militaires ou civils, volontaires ou accidentels, directs ou indirects, le risque nucléaire et radiologique est spécifique de par son impact potentiel et les dommages qu'il peut entraîner sur les biens et les populations. Dans un pays qui compte parmi les puissances nucléaires et qui dispose de 56 réacteurs en activité, ou presque, ce risque doit faire l'objet d'une attention particulière. Et si nous avons perdu une partie de notre savoir-faire en matière d'entretien des centrales, il est temps de se réassurer que nous sommes capables de gérer une telle menace. Nous souhaitons donc que la gestion de ce risque soit enseignée partout, avec les bons gestes, les bonnes pratiques et les exercices collectifs qui s'imposent. Nous aimerions, parallèlement, que soit amorcée une réflexion sur l'évolution des seuils du plan particulier d'intervention des centrales nucléaires, aujourd'hui fixé à 20

soient en quantité suffisante pour toute la population ; les réponses à nos questions sur ce point sont plutôt évasives du côté des services préfectoraux. Au vu de la politique nucléaire, à la fois civile et militaire, de notre pays, l'ajout de ces risques au plan de sensibilisation prévu par le rapport nous semble relever du bon sens Quel est l'avis de la commission ? Que le ministère

alors que le fléchage budgétaire est indispensable pour participer à l'acquisition mutualisée de moyens exceptionnels entre les Sdis. Les évolutions prévues nous semblent, de plus, sous-évaluées à la lumière des besoins capacitaires de la sécurité civile, et en particulier des Sdis, Sdis, pour faire face à l'intensification en nombre, en ampleur et en périmètre des crises, qui sont la conséquence de l'inaction climatique. Une intensification de la trajectoire pluriannuelle de la sécurité civile doit être envisagée pour accroître et moderniser les moyens matériels.

Concernant les orientations budgétaires annoncées dans le rapport annexé, nous demandons une réponse forte du Gouvernement aux besoins capacitaires de la sécurité civile, et en particulier des Sdis. Les événements climatiques extrêmes auxquels la France a été confrontée en 2022

et les présidents de conseils départementaux, de l'autre. Leur financement est tributaire de l'ensemble des collectivités territoriales, avec une participation importante des conseils départementaux, des intercommunalités et des communes,

et la politique d'asile doivent dépendre non plus du ministère de l'intérieur, mais d'un ministère dédié. La politique migratoire concerne de nombreux domaines de politiques publiques et ne doit plus être envisagée sous le seul angle sécuritaire

doublement d'effectifs en 2020, déploiement de l'opération Sentinelle, renforcement des contrôles, lutte contre le terrorisme ... Ces effets d'annonce contribuent à criminaliser l'asile et à pointer l'immigration comme un problème de sécurité nationale. pour quels résultats ? Il s'agit d'une politique vaine, coûteuse, inefficace et dangereuse, qui détourne- nous l'avons évoqué à plusieurs reprises -les agents de la police aux frontières (PAF) de leur mission de base concernant le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains.

d'accueil de l'Union européenne pour renforcer la solidarité entre ses États membres et favoriser un accueil digne des personnes exilées et réfugiées. L'amendement n° 96,

et d'un budget qui va frôler le milliard d'euros. Son développement exponentiel depuis 2015 pour faire face à l'immigration, notamment avec des agents armés, devrait se poursuivre dans une transparence exemplaire. Depuis près de deux ans,

le 28 avril dernier. Ce rapport de l'Olaf, jamais intégralement publié, ferait ressortir plusieurs accusations, notamment un non-respect des procédures, des violations des droits fondamentaux, un manque de loyauté envers l'Union européenne et une mauvaise gestion du personnel de l'agence- rien que ça Les accusations d'implication de Frontex dans de mauvais traitements, au moins de manière indirecte, remontent à plusieurs années, et se sont intensifiées depuis 2019, date à partir de laquelle les moyens de l'agence ont été décuplés. En 2019, plusieurs enquêtes menées par des médias d'investigation ont dénoncé la responsabilité de l'agence qui a toléré des maltraitances de la part de garde-frontières en Hongrie, en Grèce et en Bulgarie. Des accusations portaient également sur des agents de Frontex, lesquels auraient par exemple expulsé des mineurs non accompagnés. L'agence avait alors répondu ne pas avoir « autorité sur le comportement des polices aux frontières locales ». En octobre 2020, une nouvelle enquête de plusieurs médias rapportait l'implication d'agents de Frontex dans des refoulements illégaux de personnes cherchant refuge en mer Égée. L'enquête révélait notamment qu'un avion de Frontex avait pris des photos montrant comment un navire des garde-côtes grecs repoussait un bateau dans les eaux territoriales turques. Alors que les refoulements, pratiques illégales au regard du droit international, font désormais partie des stratégies d'éloignement de nombreux États européens- Chypre, Malte, Grèce, Lituanie, Pologne et Espagne l'implication de Frontex dans ces mauvais traitements est inacceptable. La militarisation de nos frontières a tué plus de 44 000 personnes depuis 1993 : celles-ci se sont noyées en Méditerranée, ont été abattues aux frontières, se sont suicidées dans des centres de rétention, torturées et tuées après avoir été expulsées ... Cette politique tue. Dans ce contexte, envisager une véritable intégration du corps des garde-frontières de Frontex à la gestion des frontières extérieures de la France est totalement déraisonnable. Au contraire, la France doit plaider pour une refonte complète de l'agence, qui met en oeuvre une politique aussi

Les personnes exilées font ainsi quotidiennement l'objet de pratiques illégales de l'administration française, plusieurs fois condamnée. Ce faisant, cette dernière ne respecte pas la législation en vigueur, met en oeuvre des procédures expéditives et viole les droits humains et les conventions internationales pourtant ratifiées par notre pays. Les personnes exilées sont pourchassées dans les montagnes ou sur les chemins de randonnée, sont traquées dans les bus et les trains par les forces de l'ordre. Face à cette situation, des associations travaillent des deux côtés de la frontière franco-italienne pour faire vivre la solidarité et la fraternité et ainsi redonner aux personnes exilées un peu d'espoir et de dignité. Nous devons donc réorienter notre politique migratoire et les moyens publics déployés doivent garantir le respect des droits humains fondamentaux. L'amendement 98 porte également sur l'espace Schengen. Les personnes étrangères font depuis longtemps l'objet de mesures de contrôle et de surveillance. Le fichage est devenu l'outil sans limite au service du contrôle aux frontières. L'utilisation exponentielle des fichiers destinés à identifier, catégoriser, contrôler n'est en réalité qu'un moyen supplémentaire pour éloigner et exclure. Si le fichage est utilisé pour bloquer les personnes sur leur parcours migratoire, il est aussi de plus en plus utilisé pour entraver les déplacements à l'intérieur de l'Union et l'action de militants européens qui entendent apporter leur soutien aux personnes exilées. Depuis plusieurs années, le nombre de fichiers de ce type s'est multiplié. Il en existe aujourd'hui près d'une trentaine. Leur complexité tient au fait qu'ils sont nombreux, mais également à leur superposition. De ce maillage opaque naît une certaine insécurité juridique pour les personnes visées. Parallèlement à la multiplication des fichiers de tout type et de toute nature, ce sont désormais des questions liées à leur interconnexion et à leurs failles qui sont soulevées ainsi qu'aux abus dans leur utilisation, avec notamment des risques d'atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. La justification est toujours de « protéger les citoyens européens du terrorisme international », mais il n'existe pas véritablement de données ou d'étude sur la manière dont les nouveaux registres de données biométriques et leur interconnexion peuvent contribuer à cet objectif. L'amendement vise donc à supprimer ces nouveaux fichiers et à demander la réouverture complète des frontières françaises au sein de l'espace Schengen. L'amendement n° 99, la coopération européenne en matière d'asile et d'immigration. Parmi les différentes formes d'externalisation de la politique d'immigration et d'asile menée par l'Union européenne et ses États, la sous-traitance occupe une place de choix. Cette sous-traitance s'est principalement traduite par des accords- accords de réadmission, clauses de réadmission intégrées dans des accords ou traités commerciaux, économiques ou de coopération -, en contrepartie desquels les pays concernés se voient proposer une assistance financière différents instruments de financement européens. Depuis 2002, dix-sept accords ont été conclus entre l'Union européenne et des pays non européens, auxquels s'ajoutent de nombreux accords bilatéraux mis en place par des États membres. Cette politique de sous-traitance permet à l'Union européenne et à ses États membres d'échapper à leurs obligations internationales en toute impunité et entraîne un risque d'atteinte forte au respect des droits fondamentaux, en en particulier le droit d'asile. Ces atteintes aux droits des personnes migrantes ont été largement documentées, ce qui a mis en lumière une accélération et une aggravation de ces faits depuis cinq ans. Par ailleurs, le mécanisme de Dublin a montré depuis des années son inefficacité et les injustices qu'il fait peser sur les pays du sud

est l'avis de la commission sur ces six amendements

déontologie, accueil des victimes, lutte contre les discriminations ... Ce socle a été sensiblement renforcé ces dernières années. Sa consolidation et sa pérennisation sont fondamentales. Pour poursuivre Pour poursuivre dans cette voie, les interventions gagneraient à être articulées à la réflexion plus générale sur les aptitudes, les savoir-faire et les formations relatives à la relation entre les services de police

L'alinéa 364 du rapport annexé prévoit l'allongement de la formation initiale des représentants des forces de l'ordre, de huit à douze mois, incluant un approfondissement de thématiques répondant aux enjeux clés de la police,

une réflexion des policiers sur la nature de leur mission ; en communication, y compris en tactique de médiation, de gestion des tensions ou de gestion du stress d'autrui ; sur le fonctionnement de la justice, parce qu'il n'est pas

de la formation continue, qui protégera tout d'abord le policier en lui permettant de maîtriser au mieux les outils que la société, par notre intermédiaire, se donne pour se protéger elle-même.

d'opérer un contrôle strict et régulier, non pas sur les policiers, mais sur les formations continues dans ce domaine, puisqu'elles ne sont pas systématiquement appliquées et que l'on en connaît les conséquences, qui sont, on peut le dire, Le renforcement de la formation continue d'entraînement au tir est également une revendication d'un certain nombre de syndicats de policiers, notamment la CGT Police. Aujourd'hui, trois entraînements de tir par an sont prévus et de nombreux policiers considèrent que, pour professionnaliser leur métier

Le Gouvernement affirme très clairement dans son texte d'orientation qu'il veut se rapprocher du monde de la recherche. Nous abondons totalement dans votre sens, monsieur le ministre : il faut ouvrir votre ministère à l'ensemble des champs de la recherche et des sciences.

nous appelons donc de nos voeux l'ouverture de ces formations à un certain nombre de professionnels qui pourraient les assurer- avocats, magistrats, sociologues, associations et professeurs d'université -, afin de diversifier l'apprentissage des agents présents sur le terrain, qui sont en contact permanent avec la population, et de les sensibiliser notamment aux problématiques de la délinquance des mineurs, aux problématiques économiques et sociales des habitants des quartiers et, plus généralement, aux droits humains et à la criminologie.

ne nous permet pas d'évaluer ces mutualisations puisqu'elles ne sont pas énumérées. Il est donc difficile de discuter de leur principe même. Toutefois, il nous semble important de poser un principe qui aura valeur de garde-fou : la mutualisation ne saurait se faire au détriment des besoins spécifiques des unités en fonction de leur finalité opérationnelle ou du volume horaire de ces formations. À titre d'exemple, il serait incompréhensible que les unités déployées sur le terrain comme la brigade anti-criminalité (BAC) disposent du même volume horaire de tir que les agents affectés à des tâches administratives,

insuffisant, et même dérisoire. Nous souhaitons que les agents maîtrisent correctement leurs armes, avec un volume de formation convenable. Le tir est une discipline exigeante, qui mobilise de nombreux savoir-faire dans la posture, les réflexes, la mémoire musculaire, en raison du caractère létal.

La dégradation de l'état moral, le mal-être et la souffrance des forces de l'ordre constituent le premier des constats effectués par la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure menée par le Sénat, c'est-à-dire par nous-mêmes, en 2018. Le taux de suicide anormalement élevé, supérieur de 36 % à celui de la population, constitue le révélateur de cette situation. Cet état des lieux inquiète l'ensemble des sénatrices et sénateurs, en particulier ceux de notre groupe. La lutte contre cette situation de souffrance doit être une priorité du ministère de l'intérieur. Il apparaît que l'état moral des policiers et gendarmes ne saurait être amélioré sans le concours actif des cadres de management et de commandement des personnels. À cet égard, le rapport de la commission d'enquête du Sénat soulignait le management au sein de la police nationale, jugée trop éloignée du terrain et peu à l'écoute des réalités et des difficultés des agents, contribue à la perte de sens du travail et à la démotivation des agents. Il indiquait également que les dispositifs de lutte contre les risques psychosociaux se révèlent toutefois peu efficaces si, parallèlement, les supérieurs hiérarchiques immédiats ne sont pas davantage à l'écoute de leurs subordonnés. C'est marqué au coin du bon sens dont fait toujours preuve le Sénat. Monsieur le ministre, nous ne faisons qu'expliciter votre ambition, qui rejoint la nôtre : mieux accompagner les forces de l'ordre dans leurs conditions de travail. Cela passe par un encadrement à l'écoute du mal-être, avec des outils pour aider les agents. La formation des personnels d'encadrement de la police et de la gendarmerie apparaît donc comme un levier essentiel de l'amélioration de l'état des personnels. Un supérieur hiérarchique direct en contact régulier avec ses subordonnés sera à même de les écouter et d'être attentif à leur état moral.

et que nous voyons se succéder les lois de programmation. Pour ma part, j'ai dû participer à un grand nombre de débats sur de nombreuses lois de programmation. Les lois de programmation sont belles lorsqu'on les vote.

budgétaires doivent toutefois être confirmées par les lois de finances annuelles et par la loi de programmation des finances publiques qui sera examinée très prochainement par le Sénat.

ont un rôle central dans la doctrine française de maintien de l'ordre. Elles sont des unités indispensables pour une sécurité optimale dans nos territoires, avec une mention particulière pour les CRS-MNS (maîtres-nageurs sauveteurs),

Vous avez décidé, face à cette demande, de déployer une demi-unité depuis octobre 2021, et je vous en remercie. Mais dès qu'il y a des absents ou que l'autre moitié de l'unité est déployée ailleurs, ces effectifs ne peuvent plus être présents sur notre territoire, ce qui nous laisse

La saisie d'actifs numériques introduite par l'article 3 soulève des interrogations quant à l'effectivité d'une telle mesure et son impact, à la fois sur les droits de propriété et sur le principe de proportionnalité. La jurisprudence rappelle ces droits fondamentaux,

Parmi les menaces les plus importantes, figure le, qui est un logiciel malveillant capable de bloquer les données informatiques essentielles et confidentielles de ses cibles. Une fois le forfait accompli, les pirates demandent une rançon, souvent en monnaie virtuelle, en échange d'une clé permettant de déchiffrer de nouveau ces données. Une entreprise sur cinq aurait fait l'objet d'une attaque de ce type. La gendarmerie nationale a engagé 101 000 procédures en 2020, soit une hausse de 21 %. Dans ce contexte, de nombreux professionnels de la cybersécurité, en particulier le Club des experts

Sur la forme, ils regrettent de ne pas avoir été préalablement associés à l'élaboration de cet article. Sur le fond, les acteurs du secteur estiment que cette autorisation risque d'encourager le cybercrime, voire la récidive, la multiplication d'intermédiaires douteux lors des négociations et de favoriser l'exercice d'une pression de la part des assureurs auprès de leurs clients pour les forcer à payer la rançon si celle-ci s'avère moins élevée que les frais de remédiation.

recommandé aux entreprises et aux administrations de ne jamais payer de rançon. En avril 2021, la cheffe de la section spécialisée du Parquet de Paris rappelait que la France était l'un des pays les plus attaqués.

est en rupture totale avec la doctrine préconisée par l'Anssi, ce qui aura quatre conséquences graves pour la sécurité nationale et celle de nos compatriotes. Tout d'abord, en introduisant dans le texte d'une loi française l'idée qu'une rançon peut être payée, c'est la doctrine constante de la France, selon laquelle notre pays ne paye pas de rançon, qui est remise en cause.

La France devra assumer qu'elle finance potentiellement le crime organisé, le terrorisme ou l'action offensive de gouvernements étrangers hostiles. Il y aurait aussi deux conséquences opérationnelles. Contrairement à l'objectif annoncé dans l'exposé des motifs, ce texte est un encouragement donné aux attaquants puisqu'il conforte leur modèle de rentabilité en prévoyant le financement par le paiement d'une rançon et, pratiquement, en le garantissant par une procédure d'accompagnement. La conséquence directe sera un choix préférentiel de l'attaque informatique de cibles françaises par le crime organisé, les groupes terroristes et les gouvernements étrangers hostiles. Enfin, envisager que le paiement de la rançon puisse être remboursé par les assurances est susceptible de déresponsabiliser les responsables d'entreprise. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article. La parole

souhaitent supprimer l'article 4, qui impose un dépôt de plainte pour être indemnisé par un assureur en cas de versement d'une rançon après une attaque au rançongiciel.

Nathalie Goulet -ce qui se passe sur ce sujet, et en particulier les circuits occultes de financement du terrorisme. Le paiement d'une rançon doit bien sûr rester une option de dernier recours. Lorsque la victime s'y résout, il est important, je le redis,

Cet argent sera utilisé pour attaquer encore plus de victimes. Toute disposition, quand bien même elle semblerait de bon sens, qui pourrait laisser croire que le paiement d'une rançon est quelque chose d'anodin, enverrait un terrible message.

On sait que 90 % des attaques sont rapidement signalées, ce qui facilite le travail de nos autorités compétentes afin de favoriser la récupération des données ou, dans un cas extrême, d'engager une négociation avec les cyberattaquants.

au moment de la demande de rançon, en tout cas avant le paiement. En effet, il n'est pas complètement improbable que les services de police ou les services compétents puissent détecter l'origine

monsieur le rapporteur,

Il se réfère précisément au label ExpertCyber, développé sur le site cybermalveillance.gouv.fr, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur. Le fait d'être labellisé offre une garantie supérieure de prévention du risque, avec une analyse en amont des vulnérabilités, et renforce l'ensemble du tissu entrepreneurial contre les attaques. C'est du gagnant-gagnant.

Cet article imposerait aux acteurs du secteur assurantiel de s'abstenir d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont ils savent ou présument qu'elles résultent du paiement d'une rançon exigée à la suite d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, jusqu'à ce qu'ils en aient fait la déclaration à Tracfin. Les rapporteurs de la commission ont indiqué que cette mesure était satisfaite. Néanmoins, il pourrait être soutenu que, dans le texte en vigueur, le code monétaire et financier évoque des sommes « provenant » de telles infractions alors que, dans le cadre du paiement d'une rançon, le paiement « résulte » de l'infraction. Cette précision peut peut paraître subtile, mais il s'agit d'une clarification utile, qui justifie d'adopter le présent amendement. Il nous semble que Tracfin, qui est un service de renseignement spécialisé, doit être associé pleinement à la lutte contre la criminalité économique et financière en tant qu'administration partenaire. Quel est

4G de téléphonie mobile pour transporter les communications des services de sécurité et de secours, il me semblait essentiel de renforcer la protection des infrastructures de télécommunications. Le 30 avril 2021, le ministère de l'intérieur indiquait que 174 infrastructures de télécommunications avaient été vandalisées en 2020 sur le territoire national. La prise pour cible de ces infrastructures essentielles ne s'essouffle pas, bien au contraire. Incendies de sites mobiles, sectionnements de fibres, vols de câbles ... Depuis l'été 2021, les attaques se multiplient, de sorte que le bilan de l'année 2021 a été plus lourd que celui constaté en 2020 et les six premiers mois de 2022 ont connu un record avec près de deux cents actes de malveillance recensés par la Fédération française des télécoms auprès de ses trois membres- Bouygues Telecom, Orange et SFR. Ces actes touchent désormais davantage les réseaux fixes : 159 actes ont été recensés contre 37 ayant visé les réseaux mobiles de janvier à juin 2022. L'acte le plus préoccupant a été commis dans la nuit du 27 avril 2022 : le sectionnement en plusieurs lieux du territoire des câbles de fibre optique longue distance reliant les villes de Strasbourg, Rouen, Lyon et Lille à Paris, ce qui relève du sabotage.

ce trafic que nous déplorons tous et qui transforme nos pays en une plaque tournante de produits stupéfiants avec tout ce que cela comporte comme dommages, y compris pour notre jeunesse qui s'adonne malheureusement à ce genre de pratiques.

Monsieur le ministre,